je salue notre nouveau collègue, M. Thierry Meignen, sénateur de la Seine-Saint-Denis, qui remplace M. Philippe Dallier.

Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La

Mais de quels Français parle-t-il ? Des patrons du CAC 40, ... Oh ! ... qui ont vu leur rémunération annuelle augmenter de 1,5 million d'euros en moyenne, pour atteindre près de 5,3 millions d'euros en 2021 ? Des actionnaires, qui vont voir leurs dividendes bondir à plus de 50 milliards d'euros en 2021, alors que les plans de licenciements se succèdent, surtout au sein d'entreprises qui ont reçu des aides massives de l'État Ou encore des 500 familles les plus fortunées de France, qui ont vu leur patrimoine doubler depuis le début du quinquennat ? Si c'est de ceux-là qu'a parlé Bruno Le Maire, il a raison.

Comme le dit mon ami Fabien Gay, si les salaires augmentaient comme les tarifs de l'énergie, tout le monde pourrait s'acheter un écran plat ! Ah ! Qui plus est, en cette période de rentrée scolaire, ces ménages subissent la hausse du prix des matières premières et des denrées alimentaires de première nécessité, mais aussi l'augmentation des loyers. Comme le souligne France Stratégie, les dépenses contraintes pèsent toujours plus lourd dans le budget des ménages. Monsieur le Premier ministre, améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens est une urgence. Êtes-vous prêt à augmenter significativement le SMIC, à débloquer le point d'indice des fonctionnaires et à contraindre le Medef, le Mouvement des entreprises de France, à augmenter les salaires ? Ne pensez-vous pas que les 6 % de croissance dont vous vous félicitez devraient profiter à celles et ceux qui, tout au long de cette crise sanitaire, ont fait beaucoup de sacrifices, et non pas aux plus riches, aux actionnaires ? La parole

En cette rentrée, j'ai reçu les partenaires sociaux. Madame la sénatrice, vous savez que je suis particulièrement attaché au dialogue social. Vous avez posé la question du SMIC. L'évolution de ce dernier est prévue par la loi.

notamment de l'énergie- vous avez cité en particulier l'électricité et le gaz. Nous verrons, en fonction de leur évolution, si nous devons prendre des dispositions. Et si nous devons le faire, nous le ferons.

110 millions d'euros, tel était le montant estimé et annoncé le 29 mai 2020 par Édouard Philippe, alors Premier ministre. À l'arrivée, à peine 500 000 euros ont été mobilisés, pour seulement sept communes ultramarines. Qui plus est, toutes ont dû rembourser tout ou partie de l'acompte versé en 2020, pour un montant total de 15 millions d'euros. C'est le cas des communes de Saint-Denis et de Saint-Paul à La Réunion et de Fort-de-France en Martinique, qui doivent reverser plus de 1,4 million d'euros chacune. Cela signifierait-il qu'elles n'ont pas subi de baisse de leurs recettes fiscales en 2020 ? Si, elles en ont subi, et de façon significative, mais les critères choisis pour mobiliser la clause de sauvegarde les en ont exclues

Si l'on prend l'exemple de la Guyane, mon territoire, les collectivités affichent un recul net de 15 millions d'euros, soit 5 % entre 2019 et 2020 pour les seules recettes fiscales prises en compte pour cette compensation. Avec la moyenne triennale comme référence, elles ressortent avec un surplus de 10 millions d'euros et ne sont plus éligibles à la clause de sauvegarde. Le Gouvernement a annoncé qu'il ne saurait y avoir de compensation à l'euro près ; avec ces critères, c'est en effet le cas. On voit bien qu'il n'y a pas eu de compensation et que la clause de sauvegarde n'a pas fonctionné. C'est d'autant plus pénalisant que les collectivités d'outre-mer se trouvent dans une situation financière structurellement dégradée, à l'image du contexte socio-économique et, surtout, sanitaire dans lequel elles évoluent. Veuillez conclure, mon cher collègue ! Que compte faire le Gouvernement pour y remédier ?

permettez-moi tout d'abord d'adresser mes encouragements aux Ultramarins, qui affrontent en ce moment même et depuis plusieurs semaines une vague de covid sans précédent. Les restrictions restent en vigueur dans ces territoires, afin de casser la progression de l'épidémie. Cette crise met en tension les budgets des communes qui bénéficient de clauses de sauvegarde financées par l'État. Ces mécanismes sont conçus pour aider les communes qui perdent le plus de recettes par rapport à une référence sur trois ans. J'entends votre proposition d'une référence dérogatoire pour les communes guyanaises. Nous ne l'avons pas retenue, car elle aurait créé une rupture d'égalité.

le rappelle, ce filet de sécurité se prolonge en 2021, notamment grâce à un amendement sénatorial, et s'applique également pendant ces deux années aux pertes d'octroi de mer et de taxes sur les carburants des collectivités supracommunales. le rappelle également, l'État mobilise 62 millions d'euros de subventions d'investissement supplémentaires dans le plan de relance pour les projets des communes d'outre-mer ; 8 millions d'euros la Guyane. Au-delà de la crise, je rappelle que, sur le fondement de votre rapport de 2019, nous avons engagé un rattrapage des dotations de péréquation des communes des départements d'outre-mer : alors que celui-ci était initialement prévu sur cinq ans, nous avons décidé de le mener à bien en quatre ans.

Beaucoup trop de territoires et de familles dans l'Hexagone comme en outre-mer vivent, toutes choses égales par ailleurs, les mêmes souffrances et les mêmes peines. Ils connaissent peu ou prou le même dénuement des hôpitaux, la même fatigue des soignants, la même insuffisance des effectifs et la même surdité gouvernementale. Le point commun à cette situation est donc bien la nature, la pertinence et l'efficacité de la politique sanitaire que vous conduisez. Cette quatrième vague n'est pas entrée par effraction dans nos vies. Elle est aussi la conséquence d'un sous-investissement chronique depuis des décennies dans notre système de soins et d'un manque d'anticipation manifeste dans l'Hexagone, qui a connu son acmé dans les outre-mer. Oui, votre politique porte une atteinte grave aux libertés. Elle pervertit la démocratie et installe durablement une société de contrôle. Surtout, elle ne résout en rien les carences et la désorganisation de notre système de soins. Le passe sanitaire contre lequel nous avons voté est devenu l'alpha et l'oméga de votre politique vaccinale. Il va bientôt s'appliquer à nos adolescents, avec les difficultés que l'on imagine. Soyons réalistes : les Françaises et les Français ne pourront supporter plus longtemps cette vie faite d'interdits et de restrictions. Pour notre part, sur ces travées, notre position est claire et connue de tous : c'est l'obligation vaccinale progressive, universelle et gratuite. Nous avons d'ailleurs pris une initiative de référendum d'initiative partagée pour sauver l'hôpital public et déposé une proposition de loi sur l'obligation vaccinale. Quant à vous, que comptez-vous faire pour l'avenir ? Comptez-vous maintenir encore longtemps ce passe sanitaire profondément inégalitaire et intrusif ? Quand comptez-vous enfin opter pour l'obligation vaccinale, seule mesure de nature à concilier les libertés individuelles et la protection de tous ? Quand comptez-vous enfin présenter une politique sanitaire et hospitalière repensée à l'aune de cette crise et à même de réarmer notre offre de soins ? La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.

que nous ayons décroché ne serait-ce que 5 % des crédits alloués en plus à l'hôpital au travers du Ségur de la santé : 9 milliards d'euros de hausses des salaires, 19 milliards d'euros de reprises de dette et d'investissements pour les hôpitaux, en métropole comme dans les territoires ultramarins.

Vous soulignez l'impérieuse nécessité de la vaccination. Je prends votre appel à l'obligation vaccinale comme un appel à la population guyanaise de se vacciner elle aussi. Monsieur le sénateur, on peut débattre de cette proposition, et je ne dis pas que c'est une idée saugrenue qui ne mériterait d'ailleurs pas un débat plus long que les deux minutes qui me sont accordées. que, à l'heure où je vous parle, 70 % ou 75 % de la population de Guyane ne sont pas vaccinés. J'attends donc avec impatience la proposition de loi que vous déposerez pour connaître les sanctions qui seront en vigueur dès lors que ce texte sera applicable aux 70 % de la population de Guyane qui ne sont pas vaccinés ! Encouragez-nous à vacciner les populations de métropole et d'outre-mer.

dans le contexte exceptionnel que nous traversons depuis maintenant près de dix-huit mois, le retour à une vie normale auquel nous aspirons tous passe aussi par la reprise de notre économie. L'Insee prévoit ainsi une croissance de 6,25 % pour 2021, ce qui sera malgré tout insuffisant pour compenser les trimestres de croissance perdus à cause de la pandémie. Je salue donc le plan de relance de votre gouvernement, dont l'enveloppe atteint 100 millions d'euros et qui a déjà contribué à soutenir le redémarrage de notre économie, en particulier par le pilier « cohésion des territoires », doté de 36 millions d'euros. L'investissement public est un instrument efficace de la relance. Les collectivités, qui représentent 75 % de ces investissements, sont en première ligne. Pourtant, la hausse du coût des matières premières depuis quelques mois vient lourdement grever ces investissements et,, la reprise et l'emploi. Ainsi, selon le site « commoprices.com », le prix de l'aluminium a bondi de 39 % depuis le mois de janvier dernier, celui du cuivre de 21 celui des aciers de 25 % à 80 % et celui du PVC de 52 %. Quant au bois, il devient rare et cher. Un exemple des conséquences, parmi tant d'autres : à Calamane, commune du Lot de 460 habitants située près de Cahors, le coût prévisionnel de la construction d'une école de secteur est passé en quelques mois de 1,5 million d'euros à 1,8 million d'euros, entraînant un surcoût difficile à couvrir, la commune étant à la limite de ses capacités d'emprunt. Aujourd'hui, de nombreux projets sont à l'arrêt, voire annulés, du fait de ces hausses qui se mesurent à l'échelle mondiale. Incidemment, ce sont aussi des entreprises qui se retrouvent en difficulté dans un secteur fortement pourvoyeur d'emplois. Monsieur le Premier ministre,

je veux apporter un léger correctif à ce que vous avez dit -de reconstituer le PIB détruit depuis le mois de mars 2020. Il faut travailler sur tous les leviers de la croissance ; c'est ce que mon gouvernement s'emploie à faire. faire. Parmi les sujets de la rentrée, il en est un qui est très national, si je puis dire, aux termes duquel nous créons des emplois- beaucoup, à un rythme très largement supérieur aux prévisions,

Deuxièmement, nous avons demandé aux acheteurs publics de l'État, ainsi qu'aux collectivités locales, dans le cadre des contrats de commande publique en cours d'exécution, de ne pas appliquer de pénalité lorsque des retards de livraison ou d'exécution étaient liés à des envolées de prix des matières premières ou à des pénuries d'approvisionnement.

contrats de relance et de transition écologique (CRTE) : il y en aura partout en France. Il s'agit là d'un effort massif. Nous réfléchissons, et je pourrai bientôt faire des annonces à ce sujet, monsieur le sénateur, pour aller dans le sens de votre préoccupation, à abonder

de la recherche et de l'innovation. Nous voici à la veille de la dernière rentrée universitaire du quinquennat. La mission d'information menée par le Sénat a présenté un bilan de la condition étudiante après deux années universitaires marquées par la pandémie. Elle a mis en évidence des difficultés déjà présentes, amplifiée par la crise sanitaire, notamment la précarité matérielle, l'accès au logement et à la santé. L'enquête annuelle publiée par l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, évalue la hausse du coût de la vie étudiante à plus de 2,5 % par rapport à l'an dernier et à plus de 10 % par rapport au début du quinquennat. En même temps, les aides directes ont baissé de 39 euros en moyenne par étudiant et par an, alors qu'elles avaient augmenté lors des mandats précédents. Seul un quart des étudiants reçoit une bourse, laquelle est inférieure à 200 euros pour la moitié d'entre eux. Les repas à un euro pour tous ont permis de lutter contre la précarité alimentaire, y compris pour les non-boursiers. Nous regrettons profondément la suppression de cette mesure, qui était pourtant saluée à l'unanimité. Nous souhaitons qu'elle soit réexaminée. vous avez annoncé l'embauche de 80 psychologues, 60 assistantes sociales, 1 600 référents en cité universitaire et 20 000 tuteurs. Où en est la réalisation de ces mesures à la veille de la rentrée universitaire ? Ces postes seront-ils pérennisés ? Nous arrivons au dernier projet de loi de finances du quinquennat : c'est le budget de la dernière chance pour mener une politique significative et durable à destination des étudiants. Comptez-vous mobiliser des financements pour inciter à la construction de logements en résidence universitaire ? Surtout, comptez-vous intégrer une réforme d'envergure des bourses

Vous avez raison de le dire, les étudiants ont traversé cette période avec beaucoup de résilience, de courage et de responsabilité. Ils sont aujourd'hui plus de 85 % à s'être engagés dans une procédure vaccinale, ce qui permet également cette rentrée en présentiel.

également maintenus les psychologues, car nous savons bien que la détresse psychologique que certains ont pu ressentir ne s'arrêtera pas parce que l'été est passé. L'an dernier, 77 000 consultations de psychologues ont été prises en charge pour l'ensemble des étudiants.

pour qu'ils ne se sentent pas seuls pendant la période de pandémie. Nous savons que nous aurons besoin de poursuivre toutes ces actions. Bref, madame la sénatrice, je vous rassure, le Gouvernement a été présent pour les étudiants pendant la crise. Il continuera à l'être, en espérant naturellement que cette crise s'atténue et soit bientôt derrière nous.

ont fait surgir un sujet dont on entend parler de plus en plus : quelle est la politique de gestion des cours d'eau en France et, pour être plus précis, quels sont les missions, le rôle et la place des agences de l'eau ?

des mégastructures administratives, qui se sont éloignées, pour ne pas dire déconnectées, des interlocuteurs de terrain et des problématiques locales. Elles se concentrent désormais quasi exclusivement sur la réimplantation de la biodiversité. biodiversité. C'est indispensable, mais il ne faut pas oublier en chemin tous ceux qui subissent les conséquences d'un manque d'investissement sur ces sujets. Madame la ministre, au regard de ces remarques qui remontent des territoires, pouvez-vous nous préciser les missions des agences de l'eau en la matière ? Comptez-vous avancer sur le mode de gouvernance, notamment sur le sujet très important de la composition des conseils d'administration des agences de l'eau,

Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Je m'exprime ici en tant que président du groupe d'amitié France-Afghanistan et j'associe à ma question le président Cambon et, plus largement, la majorité sénatoriale.

Le gouvernement annoncé hier laisse transparaître une ligne islamiste dure. C'est une réalité désolante, dont il convient de tirer les conséquences politiques. Les premières images du nouveau régime sont inquiétantes vis-à-vis non seulement des femmes et des activistes, mais aussi de ceux qui ont travaillé pour d'autres gouvernements. Pourtant, des signes d'ouverture avaient été donnés, notamment en direction des Devant cette situation, l'Europe et la France ne peuvent se tenir à l'écart ; les pays voisins de l'Afghanistan avancent déjà leurs pions et ont acté la prise de pouvoir des talibans. Monsieur le ministre, pour pouvoir évacuer ceux qui ne l'ont pas été, pour éviter une répression aveugle, pour protéger les vaincus du Panchir et tous les Afghans, pour préserver les acquis, notamment en matière d'éducation, et pour rétablir notre présence séculaire dans ce pays, nous nous devons de faire jouer tous les leviers. Nous n'avons évidemment aucune garantie que les talibans respecteront leurs engagements. En effet ! Toutefois, les mettre au ban de la communauté internationale nous priverait à coup sûr de tout moyen de pression et contribuerait à les rapprocher des mouvements djihadistes internationaux, à commencer par Al-Qaïda. Monsieur le ministre, une fois la poussière du chaos retombée, il vous appartiendra de définir une nouvelle stratégie vis-à-vis de l'Afghanistan. Êtes-vous, aujourd'hui, en mesure de nous en dessiner les contours ?

d'évacuation de nos ressortissants, mais aussi des Afghanes et des Afghans qui ont aidé l'armée française ou nos propres services par le passé, ou qui

préparer les conditions d'une reprise de l'économie qui, seule, pourra empêcher la crise sociale de succéder à la crise sanitaire. Aussi, je veux vous parler du tourisme, un secteur stratégique en plein essor aux Antilles, qui s'enfonce depuis mars 2020 dans une impasse, pris en tenaille entre la nécessité de maintenir des investissements indispensables à la poursuite de l'activité et l'absence durable de clientèle, sans aucune perspective d'amélioration à moyen terme. Vous avez annoncé le prolongement des dispositifs d'aide économique, comme le fonds de solidarité pour l'outre-mer. C'est une bonne chose, mais les conditions d'éligibilité font qu'un trop grand nombre d'entreprises ne peuvent y accéder. même des dispositifs d'aide à la prise en charge des coûts fixes dans l'hôtellerie et la restauration, qui excluent les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un million d'euros- soit une très large partie de nos entreprises. Le ministre des outre-mer a récemment indiqué que le plan de reconquête et de transformation du tourisme, en cours d'élaboration à l'échelon national, prendrait en considération les spécificités des territoires d'outre-mer. Je m'en réjouis, mais de quelle façon, et avec quels interlocuteurs ? Trop souvent, ces plans sont rédigés sans

Je demande une concertation étroite avec les professionnels de chaque territoire d'outre-mer, un changement de logique- tout partirait du terrain -et un plan de relance du tourisme qui nous permettrait d'attirer les investisseurs dont nous avons besoin, de rénover nos hôtels, de monter en gamme et de diversifier notre offre touristique.

Bien entendu, nous sommes attentifs à tous les trous dans la raquette qui pourraient être signalés. Nous entretenons d'ailleurs un dialogue avec les acteurs du tourisme au sein du comité de filière tourisme et avec le président de la Fédération

Résultat : une souveraineté en berne dans nombre de domaines, révélée par la crise du covid-19 et par un capital humain en déperdition. Nos talents et nos étudiants sont-ils condamnés à s'expatrier ? Que révèle l'exil des forces vives de notre pays ? pays ? La France fait-elle le choix d'être la championne de la traversée de frontières pour sa recherche et son innovation ? Pourtant, notre pays a de nombreux atouts, et la réussite de notre réindustrialisation dépend de notre capacité en recherche et en innovation. Madame la ministre, je vous adresse deux voeux, car votre ministère et la clé de voûte de notre puissance économique

En cette rentrée 2021, combien de nos bacheliers français partent au Canada, en Suisse, en Italie, aux États-Unis, en Espagne ? Je donnerai un seul exemple concret : l'École polytechnique de Lausanne compte 41 % d'étudiants français, un chiffre en hausse perpétuelle. De l'avis des spécialistes en économie, la réussite dans les filières françaises est jugée aléatoire et la formation peu épanouissante ; la peur de se perdre est au rendez-vous. Conclusion : le choix des formations étrangères s'impose. Ne dites plus que l'émigration des natifs de France est une chance pour le rayonnement national ! Elle est surtout le miroir de la faiblesse de notre attractivité pour nos jeunes talents en manque de reconnaissance. C'est une situation schizophrène pour la recherche et l'innovation, sans lesquelles, avec la formation, la puissance économique ne survit

des masters et un financement de la recherche et de l'innovation trop timide sont autant de constats du désintérêt pour les filières d'excellence et du désamour pour notre enseignement supérieur, qui manque de moyens et d'attractivité. Madame la ministre, au-delà du seul plan de relance, comment le Gouvernement entend-il prendre le virage du XXI siècle

Le Sénat s'était opposé à ce qu'il estimait être une remise en cause de la parole de l'État. De surcroît, cette baisse envoie un signal négatif pouvant décourager de futurs investissements dans le secteur si crucial des énergies renouvelables.

Heureusement, ce projet a été soumis à la concertation, et une clause de sauvegarde a été définie pour éviter que la baisse tarifaire ne conduise à des défauts de paiement. Dès lors, madame la ministre, qu'en est-il des renégociations des projets de textes d'application ? Pouvez-vous nous en dire plus sur la clause de sauvegarde ? Par ailleurs, si les économies suscitées par une telle mesure sont estimées à 500 millions d'euros par an, cette enveloppe budgétaire sera-t-elle fléchée vers le financement d'autres projets renouvelables ? La parole

toute évidence, nous devons investir des moyens considérables pour réussir la transition écologique. D'ailleurs, le Gouvernement engage ces moyens pour développer les énergies renouvelables et pour rattraper notre retard en la matière. En témoignent les 6 milliards

J'y suis particulièrement attentive, comme l'ensemble du Gouvernement, alors que nous allons prochainement adopter les textes réglementaires permettant cette révision. Comme nous nous y étions engagés, les projets de textes réglementaires ont fait l'objet d'une large consultation des acteurs, afin de

au contribuable, mais aucune des révisions ne menacera la pérennité des installations concernées. Notre ambition en matière de développement des énergies renouvelables, quant à elle, reste bien intacte. La

Les règles sanitaires locales les en empêchent, certains pays supprimant les visas de retour des expatriés qui quittent le pays. Pour ceux qui ont pris le risque de rentrer en France et qui ont été vaccinés dans leur pays d'accueil, qu'ils l'aient été avec des vaccins homologués par l'Agence européenne des médicaments ou avec des vaccins non homologués, leur vaccination n'a pas été reconnue en France. Ils n'ont eu d'autre choix que de subir des tests, la plupart du temps payants, contrairement à ce qui avait été annoncé. À la fin de l'été, alors qu'ils sont repartis dans leurs pays d'accueil, vous proposez que ceux qui auraient été vaccinés avec des vaccins listés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puissent recevoir une troisième dose, qui leur permettrait de valider leur vaccin sept jours plus tard. Avez-vous la certitude que les vaccins reçus dans les pays d'accueil et le vaccin que vous proposez pour la troisième dose sont compatibles ? De deux choses l'une : soit les vaccins utilisés, non reconnus par l'OMS et non homologués par l'Agence européenne des médicaments, sont inefficaces, voire dangereux, et vous deviez alors interdire qu'ils soient inoculés à nos compatriotes et leur fournir des vaccins agréés, soit ce n'est pas le cas, et vous devez reconnaître leur vaccination. ailleurs, dans un certain nombre de pays, dont l'Iran, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie et tant d'autres, un grand nombre de Français ne peuvent toujours pas accéder à la vaccination. Nos nombreuses interventions n'aboutissent pas. Nos compatriotes ne comprennent pas pourquoi des dispositions urgentes ne sont pas prises. Que répondez-vous à nos élus, qui sont en première ligne ?

et Républicain. Monsieur le secrétaire d'État, un an, c'est le temps dont vous disposiez pour organiser dans les meilleures conditions l'élection des six sénateurs représentant les Français établis hors de France neuf jours, c'est le temps qu'il reste avant le vote par anticipation, le 18 septembre prochain, et dix-sept jours avant le vote à l'urne, à Paris. Or certains grands électeurs, en raison des restrictions de déplacement en vigueur dans leur pays, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, ne savent toujours pas si, quand et comment ils seront en mesure de voter pour les élections sénatoriales, alors même que ce vote est obligatoire. Toutes les demandes de clarifications, voire de dérogations, sollicitées par les postes et les élus depuis des semaines sont restées lettres mortes. Mais cela semble être votre mode de gouvernance : rester sourd aux alertes et attendre la dernière minute pour réagir. Pour preuve, ce n'est que ce matin, lors d'une réunion convoquée en urgence, que vous avez consulté les parlementaires sur la tenue des élections partielles pour dix conseillers des Français de l'étranger qui n'ont pu se tenir en mai dernier, dans trois circonscriptions.

du dernier scrutin. Là encore, si vous aviez tiré les leçons du passé, vous auriez anticipé la prorogation du contrat du prestataire jusqu'à la fin de 2021. Deux mois, c'est donc le temps qu'il vous reste pour organiser ces élections partielles et celles des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE). Et pour l'instant, rien n'est prévu pour le renouvellement des membres AFE au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger. Monsieur le secrétaire d'État, ma question est simple, et votre réponse est désormais urgente : quelles instructions allez-vous envoyer aux postes, si vous ne l'avez déjà fait, pour que les grands électeurs installés en Australie et en Nouvelle-Zélande puissent voter dans quelques jours ?

les choses se préparent en bon ordre, dans le calme, en toute sérénité. Nous nous attachons, là aussi, à ce que chacun des grands électeurs puisse exprimer son vote. Vous évoquez la situation en Australie et en Nouvelle-Zélande,

autour du 7 novembre prochain, et l'AFE pourra être renouvelée vers le 5 décembre. L'Assemblée des Français de l'étranger pourra donc se réunir en toute sérénité, en bon ordre, dans le calme, et nous serons en marche pour travailler avec elle. La parole

de Haute-Provence AOP. Elle génère 9 000 emplois directs et 17 000 emplois indirects liés à l'activité touristique. Monsieur le secrétaire d'État, l'huile essentielle de lavande est un produit issu de l'agriculture française et doit le rester. Nous vous demandons que soit que soit réuni au plus tôt le comité de suivi de la réglementation Reach, et nous comptons sur votre mobilisation pleine et entière auprès de la Commission européenne pour exiger une approche spécifique, adaptée aux produits naturels et aux huiles essentielles, tout en garantissant, bien évidemment, la sécurité du consommateur et de l'environnement.

ce travail en lien avec l'ensemble des professionnels. Tel était le sens de cette première réunion organisée par Julien Denormandie ce matin. Le ministère de l'agriculture a annoncé la mise en place d'un comité interministériel d'information et de suivi,

Cela impacte directement l'ensemble des salariés et, par voie de conséquence, les allocataires. Les difficultés et dysfonctionnements informatiques s'enchaînent, perturbant ainsi le traitement des prestations familiales et des minima sociaux. sociaux. Les retards s'accumulent, avec un pic de près de 5 millions de pièces en attente. Les délais de mise en paiement de l'ensemble des prestations des allocataires sont fortement allongés. Il convient de rappeler que ces dernières représentent, pour leurs bénéficiaires, une partie importante de leurs ressources mensuelles. Cette situation n'est pas acceptable. Il est urgent que des solutions pérennes soient trouvées, particulièrement en cette période de crise sanitaire et économique. Quelles mesures immédiates seront déployées par le Gouvernement pour résoudre ce problème ? Madame la ministre, compte tenu de la gravité et de l'urgence de la situation, que comptez-vous faire

à la fois pour soutenir les agents et pour continuer les évolutions techniques du système d'information qui sont encore nécessaires. Olivier Véran, Olivier Dussopt et moi-même suivons cette situation avec beaucoup d'attention.

à chaque actualisation. C'est aussi la possibilité, demain, de rapprocher les prestations et d'aller vers un revenu universel d'activité, lequel fait toujours partie de nos projets. La parole est

Le système, à défaut d'être parfait, était au moins juste. Or, sous couvert d'une fausse égalité des chances,

le Premier ministre, la carrière doit dépendre de la valeur de chacun. Avec le système que vous allez mettre en place, ceux qui vont réussir sont ceux qui ont des relations familiales, qui font partie de réseaux occultes, tels que la franc-maçonnerie, ou qui ont des pistons politiques

l'État doit connaître ses besoins, au plus près des territoires, pour être efficace et apporter des solutions là où les Français vivent. Il s'agit donc du réarmement de l'État territorial. Deuxièmement, nous croyons aux compétences.

je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la deuxième session extraordinaire. M. le président du Sénat a reçu de M. le Président de la République communication du décret portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session Cette information sera publiée au et sur le site internet de notre assemblée. M. le président du Sénat ayant reçu communication du décret portant convocation du Parlement